La séance est reprise. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires.

interprofessions. Je considère que les avis des interprofessions sont essentiels pour compléter les dossiers d'instruction rendus par les comités techniques des Safer, afin que les décisions prises par les préfets soient les plus éclairées possible. j'ai entendu vos inquiétudes quant aux risques d'alourdir la procédure d'autorisation et de la bloquer en cas d'absence de réponse des interprofessions dans les délais impartis. Les amendements identiques n 40 rectifié et 103 visent à prévoir que les interprofessions peuvent remettre des observations écrites à tous les stades de la procédure, à la Safer, mais aussi directement au préfet si elles le souhaitent.

37 rectifié, qui tendent tous à rendre la consultation des interprofessions facultative alors que je la souhaite obligatoire. J'espère que les clarifications rédactionnelles que j'apporte, notamment pour éviter de bloquer la procédure de demande d'autorisation, répondent aux inquiétudes de leurs auteurs sur ce sujet. Pour résumer,

: La parole est à M. Joël Labbé. Cet amendement de repli tend à prévoir que le silence de l'administration vaut refus de l'autorisation d'agrandissement significatif. En l'état, le dispositif proposé établit que le silence de la Safer et de l'administration vaut accord. Compte tenu des moyens humains

dans le cadre d'un dossier d'instruction. En l'état actuel, le texte prévoit que, à défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par décret. Nous avons bien conscience qu'en France le principe est que le silence de l'administration vaut acceptation. nous savons que les dérogations sont nombreuses et nous sommes favorables au maintien de certaines d'entre elles lorsque la situation le justifie. Ce sujet sera d'ailleurs abordé demain lors de l'examen en séance de la proposition de loi visant à mettre

Cet amendement vise à supprimer les mécanismes dérogatoires prévus aux alinéas 46 à 49 permettant à un requérant de remédier à un refus de prise de contrôle par la mise en place de mesures compensatoires.

qui se révèle plus claire. Elle préserve la liberté du demandeur de l'outil de compensation choisi- la vente ou la conclusion d'un bail à long terme -, quel que soit le mode de faire valoir ou en simple qualité de propriétaire investisseur. Le statut du fermage, très protecteur, ne permet en aucun cas d'interrompre un bail rural. L'amendement

assortie d'un cahier des charges, dont le respect est encore contrôlé par les Safer. Les Safer, sociétés de droit privé, sont donc tout à la fois les instructeurs du dossier d'autorisation, les régulateurs, les « bénéficiaires » et les contrôleurs. Il s'agit là d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre

pour limiter les effets en termes de concentration, en s'engageant directement par la conclusion d'une promesse de vente ou de location par bail à long terme avec un agriculteur- un jeune agriculteur

elle préserve la liberté du demandeur de l'outil de compensation choisi- la vente ou la conclusion d'un bail long terme -, quel que soit son mode de faire valoir ou en simple qualité de propriétaire investisseur. est à M. le rapporteur. Cet amendement vise à répondre à la demande d'un certain nombre de mes collègues. Il tend à prévoir que les cessions de terres peuvent être consenties au titre des mesures compensatoires par les sociétés propriétaires, qu'elles exploitent ou non ces terres. Les

Par ailleurs, la CDOA est une instance locale rassemblant les organisations agricoles, les organismes économiques, l'État, les élus locaux, la société civile, etc. Dans cette logique, nous proposons que le préfet consulte la CDOA avant de prendre sa décision.

La commission est pourtant favorable au principe de tels remèdes constructifs : ils permettent d'autoriser la partie non excessive de l'opération tout en redistribuant une part du foncier à des jeunes et à des exploitations trop petites. C'est ce qu'on appelle du gagnant-gagnant. De telles mesures évitent en outre

le passage en comité technique des Safer sera suffisant pour que les acteurs, qui y siègent aussi pour la plupart, puissent exprimer leur position. Je rappelle que nous avons prévu qu'un compte rendu transparent de ces réunions soit transmis au préfet.

l'objet de l'amendement n° 27, auquel je suis favorable. Cet amendement me semble répondre à la demande de la plupart de mes collègues sans pour autant rendre la procédure inopérante. L'amendement n° 176 va dans le même sens, mais sa rédaction me paraît toutefois moins aboutie. L'amendement n° 101 vise lui à supprimer la possibilité de consulter la CDOA.

L'amendement n° 100 vise à supprimer la référence au SDREA. Je l'avais insérée comme garde-fou, alors que l'on prévoyait une dispense d'autorisation d'exploiter pour les projets qui auraient été instruits par cette procédure Sempastous ; mais, depuis, nous avons supprimé cette dispense.

Cabanel, pour présenter l'amendement n° 67 rectifié. Pour prendre la décision d'autoriser ou non les cessions de titres sociaux, les comités techniques des Safer seront chargés d'instruire les demandes au regard du respect des objectifs fixés à l'article L. 331-1 du code rural pour le contrôle des structures. termes du quatrième alinéa de cet article, le contrôle doit avoir pour objectif de « consolider ou maintenir des exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles Le schéma régional est donc bien mentionné parmi les critères du contrôle général des structures. C'est une bonne chose, car c'est un outil sur lequel beaucoup d'acteurs locaux s'appuient, notamment pour la mise en oeuvre d'autres politiques d'aménagement. En revanche,

bien une demande d'autorisation est considérée comme vertueuse, au regard de l'article L. 331-1 précité, qui pose d'autres conditions que je n'ai pas énumérées, soit elle ne l'est pas, et la Safer remettra au préfet un avis défavorable. La parole

On ne regardera pas de la même manière 500 hectares détenus par un seul propriétaire et non exploités et 500 hectares exploités par cinq associés et une quinzaine d'employés, faisant vivre plusieurs foyers et une filière locale.

L'accès des Safer à des informations administratives comme celles qui figurent dans le casier viticole informatisé n'est pas indispensable à l'exercice de leur mission de contrôle des transactions foncières réalisées par le marché sociétaire.

Plutôt qu'un accès illimité à de très larges données, que certains proposaient, nous avons privilégié des demandes motivées et ciblées auxquelles le préfet pourra donner suite ou non. Aussi, la

qu'elle doit rester fluide. Les Safer apprécient si l'opération de cession de titres sociaux remet en cause les objectifs généraux du contrôle de structure défini par le code rural. Elles peuvent recueillir les observations des organisations professionnelles. Il n'est pas opportun d'ouvrir la voie à une audition systématique des parties.

C'est un gage de transparence et de qualité de l'instruction, comme dans d'autres procédures administratives. L'audition des parties n'est pas obligatoire, mais, si ces dernières le demandent, elles peuvent être entendues. Un tel dispositif peut être bien cadré,

est à M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser la manière dont le préfet fixera et contrôlera le suivi des mesures compensatoires lorsque l'autorisation est conditionnée à de telles mesures. dernières seront prévues explicitement dans un cahier des charges annexé à la décision d'autorisation et feront l'objet d'un contrôle par l'autorité administrative. En cas de non-respect, le présent texte prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de l'autorisation et à la nullité de l'opération.

Les Safer ont, elles, toute l'expertise technique pour aborder cette nouvelle mission de service public, qu'elles exerceront sous le contrôle de leur commissaire du Gouvernement et de l'autorité administrative compétente.

souffrance un, deux ou trois ans après l'autorisation administrative. disposition en commission, car nous pensons qu'il faut laisser la possibilité d'opérations amiables lorsque celles-ci répondront aux critères compensatoires qui seront fixés par le préfet. En effet, en vertu de notre texte, les mesures compensatoires seront fixées par le préfet et soumises au cahier des charges réglementaires détaillé

répondant aux critères fixés par le préfet. On nous oppose parfois le manque de moyens de l'État pour contrôler le respect des conditions, mais nous parlons de moins d'une centaine de dossiers par an en France. Cet argument n'est pas recevable : charge à l'État de dédier des moyens à ce contrôle. Il me semble que le jeu en vaut la chandelle.

Le scrutin est clos.

Avant de toucher à l'autorisation d'exploiter, il faudrait conduire un travail de fond en évaluant ses résultats actuels, en examinant comment elle est menée par les services déconcentrés et en comparant diverses pistes de réforme.

amendements du Gouvernement,

dès lors que la Safer instruit le dossier de demande pour le compte de la préfecture, elle ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts. En outre, son rôle est de protéger les terres agricoles et elle intervient à 90 % à l'amiable et non en préemption. La parole est à Mme

ou des titres sociaux concernant les sociétés dont elles auront pu instruire les demandes d'autorisation, même si, comme cela a été rappelé plusieurs fois dans cet hémicycle, le dispositif initial écartait tout risque de conflit d'intérêts : c'est l'autorité administrative qui décide, en toute circonstance, de la nécessité de mettre en place des mesures compensatoires

qui met à mal les outils existants au lieu de les renforcer. En gelant les moyens d'intervention des Safer, on risque de les fragiliser fortement et ainsi de menacer leurs missions d'intérêt public, notamment pour le renouvellement des générations. Cette mesure constituerait également une voie évidente de contournement : en passant par le nouveau dispositif de contrôle, on est à l'abri des dispositifs de régulation confiés aux Safer pour neuf ans. On peut imaginer qu'un déclarant dépose un jour une demande d'autorisation pour la réalisation d'une opération quasi insignifiante pour échapper ensuite au contrôle sur une opération plus problématique.

M. Christian Klinger. Cet amendement vise à améliorer le contrôle du respect des engagements pris par les parties aux opérations sociétaires qui ont été autorisées sous condition, en permettant à la Safer d'intervenir sur les terrains concernés en appui du préfet. du texte de la commission, la Safer ne peut intervenir, pour une durée de neuf ans, sur les biens des sociétés dont elle a instruit les opérations dans le cadre de la procédure de contrôle créée par cette proposition de loi. dans le cas où des engagements ont été pris auprès du préfet par les parties à l'opération- par exemple pour céder une partie du terrain ou le mettre à bail à un agriculteur souhaitant s'installer -, il faut s'assurer que l'ensemble des engagements seront tenus pour toute la durée prévue.

insuffisamment ou lorsque le cahier des charges fixé par le préfet n'est pas respecté, nous proposons donc que la Safer puisse intervenir sur les terrains concernés, par exemple en faisant usage d'une préemption dès la prochaine cession. Rappelons que le préfet peut aussi prendre des sanctions administratives, allant d'une mise en demeure ou d'une amende au retrait de l'autorisation et à l'action en nullité.

les demandeurs de soupçons de conflits d'intérêts, alors que le texte leur donne de nouveaux pouvoirs d'instruction très étendus, qui dépassent de loin leur rôle actuel. La Safer instruirait le dossier et, nous l'imaginons bien, suggérerait au préfet et au demandeur des mesures compensatoires, qui se traduiraient ensuite par des ventes à leur bénéfice. Certes, l'objectif serait d'installer des jeunes ou de consolider des exploitations, mais rien n'empêche de le faire à l'amiable.

Ne faisons pas croire que nous amputons le pouvoir ordinaire de régulation des Safer ! La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 112 rectifié, qui vise à lever l'interdiction faite aux Safer en cas de non-respect par le demandeur des conditions fixées par l'autorisation. Les Safer pourront, le cas échéant, préempter le terrain ou acquérir des parts de la société, pour les réattribuer à des jeunes, par exemple. Pour ces raisons, moyennant les garde-fous nécessaires et tout en soulignant l'amélioration bienvenue apportée par l'amendement n° 112 rectifié, je souhaite maintenir le texte de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

sous forme de comptes rendus. La composition des comités techniques dépendant du cadre réglementaire, il n'est pas utile de l'inscrire dans la loi. de même pour la publicité des travaux de ces comités, dont il convient de rappeler que les débats ne sont pas publics, que les avis qu'ils sont amenés à rendre sont purement consultatifs et que les décisions qui sont prises à la suite de leurs avis sont motivées et publiées.

notre débat. L'objectif est d'améliorer l'impartialité et la transparence des avis rendus par les Safer et de bien exclure les membres des comités techniques des réunions et des avis sur des affaires pour lesquelles les Safer peuvent avoir à se prononcer. Il s'agit d'une question de transparence. Cet amendement me semble de bon sens.

Il me semble normal et nécessaire qu'un comité doté d'un tel rôle ait une composition minimale garantie par la loi, pour assurer une égalité de traitement dans les territoires. L'amendement n° 5 rectifié a quant à lui pour objet d'exiger une déclaration d'intérêts pour tous les membres du comité technique.

contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle avait voulu étendre le droit de préemption des Safer à une cession de biens immobiliers agricoles importants logés dans une société dédiée.

qui opère une extension démesurée des capacités des Safer. Il est essentiel, selon nous, que toute nouvelle arrivée d'un associé dans une société soit pleinement consentie par les autres exploitants, pour que cela fonctionne. C'est une question non pas technique, monsieur le ministre, mais politique ! L'article donne à la Safer le pouvoir d'imposer, après mise en concurrence des parts, un nouvel associé dans une exploitation existante. L'initiative de la vente viendrait bien des associés, mais ceux-ci n'auraient pas leur mot à dire dans le choix du nouvel exploitant. Il y a donc là un risque constitutionnel. En outre, cette nouvelle capacité n'est plus nécessaire, car nous avons supprimé l'intervention obligatoire des Safer dans toute mesure compensatoire à l'article 1, au profit d'un cahier des charges préfectoral. J'insiste sur ce point

qui figurent dans le casier viticole informatisé

et, d'autre part, de ne pas limiter cet accès pour les besoins de l'instruction des seuls dossiers portant sur des opérations sociétaires. La condition imposée par cet alinéa serait matériellement très difficile, voire presque impossible, à remplir ou à mettre en oeuvre dans le délai normal d'instruction d'un dossier.

Les Safer considèrent à juste titre que cela introduit manifestement un obstacle au bon exercice de leur mission, ce qui ne leur permettra pas de conduire efficacement l'instruction des dossiers. En conséquence, cela empêchera l'autorité administrative compétente d'être suffisamment éclairée dans sa prise de décision.

Cette évolution vise à éviter les pressions, notamment financières, qui peuvent exister et qui conduisent à éliminer des demandeurs prioritaires, particulièrement des candidats à l'installation en agriculture. Dans un souci de cohérence et d'efficacité des politiques foncières, il est nécessaire d'adapter les outils de contrôle de l'accès au foncier agricole, en ouvrant à l'autorité préfectorale la possibilité de refuser une autorisation d'exploiter dès lors que celle-ci est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations du schéma directeur régional des structures agricoles.

ou une concentration excessive de l'exploitation correspond à la philosophie du texte. Il s'agit de fournir aux préfets un levier supplémentaire en faveur de l'objectif d'installation des jeunes agriculteurs.

Nous cherchons tous à préserver avant tout l'activité agricole en France face aux risques de déprise. Or cet article permettait aux préfets de refuser une autorisation à un exploitant, alors même qu'aucun autre exploitant ne serait intéressé par la reprise de l'exploitation

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

Qu'il s'agisse des bâtiments, de la valeur ajoutée du terrain ou de bien d'autres aspects, il est essentiel de mieux définir le foncier et ses différentes parts, de manière méthodique et approfondie.

Cette proposition de loi intervient après un certain nombre de faits divers qui se sont déroulés il y a cinq à six ans. Les Safer ont réussi à démontrer qu'il existait encore des pans du droit rural qui leur échappaient

Nous espérons que, après le temps des débats, viendra celui du compromis en commission mixte paritaire, car, comme l'indique l'intitulé de cette proposition de loi, il y a urgence. Nous voulons avancer. Nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi.

Les discussions ont été riches et quelquefois bouillonnantes, sur un sujet particulièrement technique. Il fallait nous saisir de ce texte que nous savions essentiel et prendre en compte l'intérêt général.

L'outil sociétaire a été identifié comme un instrument privilégié d'acquisition- certains diraient « d'accaparement » -des terres agricoles. Quoi qu'il en soit, ce modèle s'est beaucoup développé dans le monde agricole, car il présente des avantages. Il protège le patrimoine personnel en le séparant du patrimoine professionnel, il permet de dissocier les types d'imposition et il facilite la reprise des exploitations.

Les outils actuels ne permettent qu'un contrôle limité, qui ne s'exerce pas sur les cessions partielles de parts de sociétés agricoles. Le Sénat a choisi de maintenir ce dispositif dans ses grandes lignes et de le rééquilibrer. recentré sur la lutte contre la concentration excessive et l'accaparement des terres agricoles. Nous avons délimité le rôle de chaque acteur, ajusté certains paramètres du contrôle et clarifié la procédure. Nous nous sommes aussi attachés à trouver un compromis entre la préservation des libertés constitutionnelles

le Sénat dans ses travaux : territorialiser pour rapprocher la prise de décision du terrain ; recentrer le dispositif pour qu'il réponde mieux aux objectifs affichés, à savoir lutter contre l'accaparement des terres agricoles et faciliter l'installation des jeunes agriculteurs

qui ont constitué, génération après génération, année après année, sacrifice après sacrifice, un capital d'exploitation,